le 27 septembre 2024, un étudiant de l’université Paris Panthéon Assas a été violemment agressé par des militants d’extrême droite aux portes de cet établissement. Il sortira de l’hôpital avec huit jours d’incapacité totale de travail (ITT). Cette agression n’est pas un acte isolé. Depuis plusieurs années maintenant, la violence de l’extrême droite gagne du terrain dans les établissements d’enseignement supérieur. Le sentiment d’impunité est total au sein de ces collectifs. La banalisation des actes et propos racistes, homophobes et sexistes rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Paris, Besançon, Reims, Bordeaux, Lorient, etc. les signalements se multiplient face à la recrudescence de la création de collectifs ouvertement radicaux, qui n’hésitent pas à s’afficher avec des symboles néofascistes et à relayer sur les réseaux sociaux des actions violentes et intimidantes. Le climat politique est particulièrement délétère et je souhaite alerter le Gouvernement sur la dangerosité de ces groupes d’extrême droite. En effet, monsieur le ministre, vous ne semblez pas avoir pris conscience de cette recrudescence. Volontairement ou non, votre absence de prise de parole sur ce sujet est extrêmement problématique. Les étudiantes et étudiants, quels que soient leur origine sociale, leur orientation sexuelle ou leur genre, doivent être protégés et doivent se sentir en sécurité dans la poursuite de leurs études. Nous avons un combat à mener pour une connaissance plus précise de ce phénomène et pour le déploiement de mesures de prévention ciblées et de moyens spécifiques, afin de lutter contre la résurgence de l’extrême droite dans les établissements d’enseignement supérieur. Quelles actions prévoyez vous de conduire à cet égard ? Ce combat doit être mené en front commun et républicain.

ma position est constante et ne saurait s’écarter des principes de notre démocratie et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont l’article 11 dispose : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Tout est dit. L’université est, par essence, le lieu où la liberté d’expression est garantie, dans un cadre délibératif, c’est à dire permettant le débat contradictoire. Je l’assume, l’université est libérale, au sens classique des libertés garanties : liberté académique, liberté d’expression, liberté d’enseigner et, bien entendu, liberté d’étudier. Mais je ne tolère aucune atteinte tant aux aux personnes qu’aux biens. Les auteurs de violences doivent être poursuivis et sanctionnés pénalement et administrativement. Que les choses soient claires, aucune violence n’est tolérable, d’où qu’elle vienne. La circulaire du 4 octobre 2024 a visé à rappeler aux gouvernances des établissements les pouvoirs à leur disposition pour s’assurer que chacun puisse étudier et enseigner sereinement. Chaque fois que la situation l’exigera, les chefs d’établissement pourront saisir le procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, et je soutiendrai systématiquement ces actions. Je l’ai par ailleurs précisé dans ma feuille de route, le ministère diffusera

des événements signalés, tels que ceux auxquels vous venez de faire référence. Le dispositif ministériel de veille, d’alerte et de signalement des événements graves est opérationnel de façon continue depuis septembre 2023. Au sein de chaque établissement, les FSD diffusent une

Monsieur le ministre, à quelques semaines du, comme on l’appelle en bon français, je souhaite attirer votre attention sur les accidents liés à l’alcool et aux stupéfiants lors des soirées étudiantes organisées dans les locaux des établissements d’enseignement supérieur ou universitaire. La diffusion du modèle américain des soirées de promotion étudiantes ou la radicalisation des soirées d’intégration dans les écoles supérieures ont entraîné au fil des années de nombreux accidents dramatiques, voire tragiques, qui ont coûté la vie à de jeunes adultes. le deuil des parents, des sœurs, des frères, des camarades et des établissements entiers. Ce fut malheureusement le cas dans notre département de Saône et Loire. Ces événements qui se déroulent soit dans le cadre strict des locaux scolaires, soit aux abords ou à la sortie de ces soirées, sont bien souvent la conséquence de jeux de boisson et de rituels alcoolisés, possiblement accompagnés d’une consommation de drogue à l’origine de ces drames. Aussi, compte tenu du caractère institutionnel ou conventionné des établissements scolaires ou universitaires organisateurs, et au vu des drames occasionnés, l’État ne saurait se désintéresser du sujet. Des mesures concrètes doivent être mises en place pour que les organisateurs de ces soirées préviennent les conduites à risques, afin d’assurer la sécurité des étudiants. C’est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir m’indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que ces accidents soient évités et pour que des vies soient épargnées.

contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Le simple fait de promouvoir et d’organiser des soirées où tout excès est encouragé est puni par la loi. Particulièrement sensible à cette question, j’agis avec mes services de deux manières : les signalements pour punir les auteurs et accompagner les victimes, d’une part,

Je vous assure de ma grande réactivité devant de telles dérives. En effet, outre la mise en danger de la jeune personne promise à un bel avenir, à laquelle vous faisiez référence à l’instant, je ne peux accepter que ces moments d’excès d’alcool, voire de drogue, soient susceptibles de donner et violences sexuelles. Or il s’agit aussi, il faut le dire, d’une réalité. C’est pourquoi le ministère de l’enseignement supérieur conduit, depuis deux ans, la campagne de communication intitulée « Sans oui, c’est interdit », centrée sur le

». Ils déclarent avoir subi un bizutage incluant pratiques humiliantes, comportements dégradants, voire actes sexuels non consentis. Malgré son caractère illégal depuis 1998, le bizutage continue de bénéficier d’une tolérance liée à la persistance de certaines traditions, comme à la mise en œuvre de rapports de pouvoir entre anciens et nouveaux, qu’une interdiction formelle ne parvient pas à endiguer. Les week ends d’intégration sont totalement inclus dans l’aspect « business » de nombreuses grandes écoles, lorsqu’ils ne participent pas de leur réputation positive. Leur organisation hors les murs des établissements participe de cette culture et de la persistance de ces conséquences. La responsabilité des établissements et de leurs chefs est en tout état de cause engagée. Les règlements intérieurs doivent s’appliquer et les procédures disciplinaires s’enclencher, y compris quand les faits ont lieu à l’extérieur. Une procédure pénale est toujours possible. Certains rites étudiants, même sous une forme parfois édulcorée, demeurent le paravent ponctuel d’abus inacceptables mettant en cause la sécurité et la santé des étudiants. Monsieur le ministre, quelles dispositions entendez vous prendre afin de mettre un terme aux excès constatés afin de protéger, davantage et encore mieux, les étudiants.

ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » Il existe au sein de chaque établissement un dispositif de signalement, qui rend effectifs à la fois le suivi et la sanction de ces actes lorsque c’est nécessaire. À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre dernier, le ministère a adressé à l’ensemble des présidents d’université et aux chefs d’établissement un guide opérationnel pour les accompagner dans la mise en œuvre et le suivi de ces dispositifs. Par ailleurs, pour les victimes, la Coordination nationale d’accompagnement des étudiantes et des étudiants (Cnaé), créée en 2023, assure un suivi et, bien entendu, une orientation nécessaire. Pour éviter que ne surviennent de telles situations, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a aussi déployé un ensemble de mesures visant à prévenir les actes de bizutage et les violences sexistes et sexuelles.

de l’éducation nationale. Monsieur le ministre, l’éducation nationale est le socle de notre République. Elle est garante de l’égalité des droits et des chances pour tous les élèves, quel que soit leur lieu de résidence. Or l’annonce du projet de budget pour 2025 suscite à cet égard une vive inquiétude dans nos territoires, notamment en milieu rural. Ces territoires risquent d’être de nouveau les premières victimes d’une baisse massive de moyens par la suppression de 4 000 postes d’enseignant, dont 3 815 dans le premier degré. À titre d’exemple, dans le département dont je suis élu, le Cher, 31 classes ont déjà fermé l’an dernier et 19 postes d’enseignant ont été supprimés. Ces chiffres, que je trouve alarmants, traduisent une tendance lourde à la dégradation de l’encadrement pédagogique, qui affecte directement les élèves et creuse les inégalités territoriales. En zone rurale, nous assistons à la fermeture d’écoles, qui sont pourtant des lieux de vie essentiels. En zone urbaine, les classes sont surchargées, ce qui complique les efforts des enseignants pour offrir à chaque élève une attention adaptée.

Cette vision éclaire notre devoir collectif : l’instruction de nos enfants est un honneur pour notre pays. Que comptez vous faire pour protéger cet honneur, en particulier dans nos zones rurales qui, année après année, se sentent reléguées ? Quelle est votre stratégie pour garantir

Compte tenu de cette baisse très importante, on constate une amélioration du taux d’encadrement, exprimé en nombre d’élèves par classe : en 2024, l’enseignement primaire public accueille

avec les élus locaux – du moins faut il l’espérer –, et qu’ils ont lieu sur la base d’une appréciation fine et objective de la situation de chaque école et des spécificités des territoires. La répartition des moyens dans le premier degré tient notamment compte du caractère plus ou moins rural, à la fois, de chaque académie, de chaque département, puis de chaque circonscription, et même de chaque école. Pour mieux répondre aux préoccupations exprimées par les élus locaux, en 2024, le dialogue et la coordination ont été renforcés en amont des fameux conseils départementaux de l’éducation nationale dans le cadre de l’Observatoire des dynamiques rurales. Des réponses adaptées aux territoires ruraux ont été élaborées au cours des dernières années, notamment l’allocation progressive des moyens ou encore le dispositif des territoires éducatifs ruraux, qui constituent une avancée. S’agissant plus particulièrement du département du Cher, dans un contexte de forte baisse démographique, les taux d’encadrement se sont nettement et constamment améliorés. Ainsi, le nombre d’élèves par classe y était de 20,6 à la rentrée 2024,

offrir à chaque élève en situation de handicap les conditions nécessaires à sa réussite scolaire et à son épanouissement personnel. Or de nombreux témoignages montrent que ce droit, pourtant essentiel, n’est pas toujours assuré.

changement en cours d’année. Nous saluons collectivement le travail remarquable des AESH. Je veux naturellement leur rendre hommage, car ils jouent un rôle clé dans la vie de ces enfants. Chaque nouvel accompagnant devient pour l’enfant un repère essentiel. À ce titre, il est d’autant plus crucial de garantir la stabilité de la présence des AESH auprès de ceux qu’ils accompagnent. Pourtant, les ruptures d’accompagnement s’enchaînent, ébranlent la confiance de ces élèves et rendent leur inclusion de plus en plus incertaine. Notre pays compte des centaines de Paul Axel, qui subissent chaque année les mêmes désagréments. de l’éducation nationale compte t il mettre en œuvre pour garantir aux enfants en situation de handicap la stabilité de leurs accompagnants, condition indispensable pour que leur inclusion soit effective ? Envisagez vous de prendre des mesures pour renforcer le dialogue entre les équipes éducatives et les familles, afin de sécuriser le parcours scolaire de ces élèves

essentiel de notre République. Nous mettons tout en œuvre pour assurer une scolarité de qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée, quels que soient leurs besoins éducatifs particuliers, et avec l’ensemble des équipes pédagogiques, auxquelles je veux ici rendre hommage. À la rentrée 2024, 519 000 élèves en situation de handicap qui ont été scolarisés, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. En cette rentrée scolaire, 332 000 élèves sont notifiés pour un accompagnement humain, soit une augmentation de 28 000 par rapport à l’année précédente. Nous développons des mesures pour renforcer l’accessibilité des apprentissages, comme le matériel pédagogique adapté, mais aussi le nombre d’accompagnants des élèves en situation de handicap, qui participent quotidiennement à construire une école toujours plus inclusive. Pour rappel, au niveau national, 15 000 postes d’AESH ont été créés en quatre ans, dont 3 000 à la rentrée 2024. Ces moyens importants sont l’un des leviers permettant de garantir la continuité de l’accompagnement humain, quels que soient les projets d’évolution de nos personnels – vous avez raison d’insister sur ces aspects. La loi du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne est un autre levier pour assurer la continuité de l’accompagnement des élèves. L’attention portée aux familles est un objectif fondamental pour garantir un cadre de confiance réciproque et assurer une scolarisation réussie pour tous. C’est pourquoi les pôles d’appui à la scolarité, dispositif de proximité issu de la dernière Conférence nationale du handicap (CNH), ont également été créés. Leur mise en œuvre dans quatre départements préfigurateurs a vocation à permettre de meilleures répartitions et attributions des AESH, et à répondre plus rapidement aux besoins des élèves, en sollicitant le cas échéant les services médico sociaux. Vous avez raison, il faut que tout cela aille encore plus vite. En tout cas, le Gouvernement s’y emploie. La parole

nombre de collectivités se voient dans l’obligation d’abandonner des projets en raison de contraintes trop importantes qui impactent très fortement leurs budgets. Ces exigences, parfois ubuesques, sont incomprises. Assurément, les élus n’ont pas l’intention de dénaturer leur commune, et ce sont eux qui connaissent le mieux leur patrimoine. Leur souhait est de travailler en collaboration avec les architectes afin de trouver un consensus qui prenne en compte les besoins architecturaux, les capacités financières de la commune, mais également le cadre global du projet. dans certains cas, les exigences purement subjectives des ABF ne sont pas acceptables. Dans le contexte où se trouvent nos collectivités, je souhaiterais savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour diminuer les contraintes sur les projets locaux,

Les architectes des bâtiments de France sont chargés de la conservation des sites protégés en raison de leur intérêt patrimonial, tels que les abords des monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables classés au titre du code du patrimoine. Ces espaces contribuent au rayonnement culturel et à l’attractivité touristique et économique de notre pays. Or, sans le contrôle des ABF, ils ne seraient sans doute pas protégés ; c’est alors le régime commun du droit de l’urbanisme qui s’appliquerait. Je rappelle que l’avis de l’ABF est toujours rendu au cas par cas, en fonction de chaque projet et des enjeux locaux de préservation du patrimoine,

seuls 7 % font l’objet d’un avis défavorable. Un premier projet refusé est par ailleurs souvent suivi d’un nouveau projet qui, lui, sera accepté. Enfin, une procédure d’appel existe en cas de désaccord entre le porteur du projet et l’autorité compétente. En l’occurrence, les élus peuvent

durant les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024. Ces Jeux ont été, rappelons le, une véritable réussite pour Paris et pour la France. Ce succès a été possible grâce au travail remarquable des forces de l’ordre et des militaires, qui ont assuré une sécurisation exceptionnelle des sites olympiques et des zones sensibles, sous l’autorité de la préfecture de police et du gouverneur militaire de Paris. Je tiens d’ailleurs à leur rendre hommage. Cependant, de nombreux commerçants parisiens ont été directement et négativement affectés par les dispositifs de sécurité déployés pendant plusieurs semaines, notamment dans le XVII arrondissement Je peux citer, par exemple, les commerçants de l’avenue de la Grande Armée, de l’avenue de Wagram ou encore de la place Charles de Gaulle. Le 12 juin dernier, le préfet Michel Cadot, délégué interministériel aux JOP, avait annoncé la création d’une commission nationale pour indemniser les établissements économiquement affectés par les restrictions liées aux Jeux. Or cette commission ne s’est toujours pas réunie alors que les commerçants subissent, plus que jamais, les conséquences économiques de ces restrictions, qui mettent en péril leurs activités et leur avenir. Madame la ministre, pouvez vous confirmer la création de de cette commission, et nous en préciser ses modalités ? De plus, pouvez vous nous assurer que les commerçants concernés pourront bénéficier d’un mécanisme juste et équitable d’indemnisation ?

des consommateurs. Clauses illicites contraires au code de la consommation, clauses présumées abusives sur les modalités de réservation des places, communications mensongères, allégations trompeuses : ces pratiques nombreuses portent préjudice aux familles.

pourquoi la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), chargée du contrôle des grandes entreprises, n’a t elle pas été sollicitée ? Pourquoi le nouveau conseil d’évaluation des fraudes, dédié à l’évaluation du montant des fraudes aux aides publiques, ne s’est il pas vu confier une mission sur les grands groupes de crèches privés ? En attendant, en octobre, les salariés de People & Baby n’ont touché qu’un acompte

de la sécurité sociale pour 2025 –, permettra de garantir un accueil de qualité pour tous les enfants et leurs familles. Ce service public sera accompagné d’un système de contrôle en lien avec le ministère. À plus long terme, le Gouvernement a pour objectif de réformer le mode de financement des crèches pour aller vers un système plus juste et davantage centré sur la qualité de l’accueil. Nous devons définir les conditions d’évolution de l’ensemble des modes de financement, qu’il s’agisse de la prestation de service unique, du financement des microcrèches ou des conditions d’investissement.

Son objectif est de renforcer la structure financière de l’entreprise et de permettre le financement de sa refondation. Cette procédure judiciaire, qui prendra entre deux et quatre mois, devrait permettre au groupe de restructurer son passif, d’obtenir de nouveaux financements et de se relancer sur des bases saines.

Alors que les enjeux sont cruciaux pour la modernisation de notre pays et que les efforts doivent être intensifiés, les orientations budgétaires actuelles prévoient une diminution des autorisations d’engagement et des crédits de paiement alloués à ce plan. Cela risque de compromettre la réalisation des objectifs d’accès à la fibre pour 2025, notamment dans les zones d’initiative publique lorsque ces raccordements sont qualifiés de complexes.

Madame la ministre, de quelle façon le Gouvernement entend il garantir le financement et le respect des délais pour le déploiement de la fibre dans tous les territoires ? La parole

La réussite de ce plan est d’ailleurs le fruit d’une alliance entre l’État, les collectivités, que je salue, et les opérateurs privés. Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, le soutien de l’État depuis 2010 s’élève à 3,57 milliards d’euros. Pour le soutien aux projets de réseaux d’initiative publique (RIP) des collectivités, l’État a mobilisé, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), plus de 2,24 milliards d’euros de subventions.

En Mayenne, le projet d’investissement Niagara du groupe LDC, d’un montant de plus de 150 millions d’euros, vise à renforcer les sites de Lassay les Châteaux et de Laval. Ce projet est crucial pour la résilience et la compétitivité de notre secteur avicole. Il est en effet important de permettre aux Français de consommer du poulet né, élevé et préparé en France. Initialement, le projet Niagara a été reconnu comme l’un des dix projets prioritaires au niveau national, ce qui souligne son importance stratégique. Cependant, les porteurs de ce projet ont récemment reçu un retour négatif de Bpifrance à leur demande d’accompagnement dans le cadre du plan France 2030, et ce sans information préalable. Les critères ayant conduit à ce refus ne sont pas clairs. Malgré de multiples demandes de clarification durant la période d’instruction, Bpifrance n’a pas fourni de réponses permettant d’ajuster le dossier. Cette décision intervient alors que les agriculteurs sont mobilisés face aux défis posés par les accords potentiels entre l’Union européenne et le Mercosur, qui menacent notre souveraineté alimentaire. Madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement envisage t il de prendre pour garantir l’accompagnement transparent et équitable des projets stratégiques ? Peut on s’attendre à un renforcement du soutien à nos producteurs locaux face à la concurrence internationale,

Le projet Niagara vise à augmenter considérablement les volumes de viande de poulet destinés aux débouchés en dehors des grandes et moyennes surfaces (GMS). Il représente un investissement important pour le groupe, dans un contexte de tensions sur les prix et de risques sanitaires accrus.

d’obtenir un soutien public pour la réalisation de ce projet d’ampleur. Selon la procédure d’instruction, le dossier a été étudié par les services de Bpifrance, opérateur de ce dispositif, les services de l’État et des experts indépendants.

Par ailleurs, la capacité de la France à verser des aides aux entreprises est encadrée à l’échelon européen par des régimes d’aides d’État. L’analyse du dossier de demande d’aide a révélé qu’il n’était pas possible d’aider ce projet au regard des régimes

Si cette aide est la bienvenue, en particulier pour de nombreuses communes rurales de mon territoire, engagées dans une grande diversité de projets, la répartition des montants engagés par département interroge.

de la carte postale de la riviera azuréenne – certes urbanisée –, comporte de nombreuses petites communes rurales. En effet, à titre d’exemple, dans un département comparable du littoral méditerranéen que je ne citerai pas,

fait le choix de maintenir cette dotation à un niveau élevé, avec une enveloppe de 1 milliard d’euros pour 2025. Comme vous le rappelez, l’enveloppe de DETR a été fixée pour les Alpes Maritimes à 3,01 millions d’euros en 2024.

à la moyenne nationale, cela résulte de la combinaison des critères fixés à l’article L. 2334 35 du code général des collectivités locales, à savoir non seulement la population, mais également la densité et le potentiel des communes. Le législateur a, en effet, choisi de retenir des critères de répartition qui permettent de concentrer les moyens financiers de la DETR sur les départements les plus ruraux, dont les ressources sont comparativement souvent beaucoup plus faibles. Ainsi, et c’est heureux, les Alpes Maritimes regroupent des collectivités au potentiel financier plus élevé que la moyenne, qui se caractérisent

a sollicité la réorientation d’une petite partie des aides, à budget constant, afin de permettre l’importation d’aliments pour bétail sans organismes génétiquement modifiés (OGM), contribuant ainsi à la production d’une viande exempte d’OGM par les producteurs locaux. Cette requête a fait l’objet d’une concertation locale et a abouti à un avis favorable du comité d’orientation stratégique et de développement agricole (Cosda), le 27 septembre 2024. été validée à l’unanimité par la collectivité territoriale de Martinique (CTM) lors de sa délibération du 4 octobre 2024, puis par les services du ministère de l’agriculture et

il semble que cette modification n’aurait pas été transmise à la Commission européenne. Aussi, je souhaite savoir quand cette décision validée à tous les niveaux, prise dans l’intérêt des Martiniquais et visant à garantir une production de viande saine, pourra être dûment transmise aux autorités européennes. Le cas échéant,

Il s’agit d’un enjeu majeur de santé publique, qui rend nécessaire une réponse rapide et claire, afin de garantir aux producteurs et aux consommateurs martiniquais un cadre sécurisé et conforme aux objectifs fixés collectivement.

Nous disposons en effet du régime spécifique d’approvisionnement (RSA) dans le cadre du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité. Il permet de subventionner une part significative

ainsi que pour l’entretien des kilomètres de pistes de défense des forêts contre l’incendie, les forestiers sapeurs, classés comme agents sédentaires de la fonction publique, demandent légitimement à être reconnus comme relevant de la catégorie active, à l’instar de leurs collègues sapeurs pompiers professionnels ou d’autres emplois de service public comme les infirmiers, les sages femmes ou les assistantes sociales. Ce changement statutaire tant attendu par les intéressés entraînerait une reconnaissance des risques et de la pénibilité de leur travail ainsi que l’octroi de primes, justifiées au regard des dangers encourus

déterminant des forestiers sapeurs dans la politique de prévention et de sauvegarde de la biodiversité ainsi que dans l’appui qu’ils apportent aux missions héliportées

phénomènes naturels, constat particulièrement vrai en Dordogne face au retrait gonflement des argiles. Il est urgent de réformer les critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, afin de mieux répondre aux attentes des territoires. deux arrêtés ministériels publiés en 2024, la totalité des demandes de 170 communes de Dordogne au titre des « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » pour l’année 2023 Ces critères, complètement déconnectés des réalités du terrain, ne répondent pas aux attentes des maires et des habitants touchés. Les sinistrés, qui constatent quotidiennement l’aggravation des dégâts sur leurs bâtiments, ressentent ces décisions comme une profonde injustice.

proviennent exclusivement de Météo France. Elles ne sont pas systématiquement accessibles ni même précises, alors qu’elles justifient les rejets. Il est urgent de modifier la méthodologie en intégrant les données locales, notamment celles que fournissent les chambres d’agriculture

offrent une vision bien plus fine des phénomènes climatiques que celles de Météo France. Elles sont aussi plus accessibles, grâce à des plateformes partagées avec les techniciens et avec les agriculteurs. Monsieur le secrétaire d’État, allez vous enfin prendre en compte ces données locales dans les critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ? Cette démarche permettrait de garantir des décisions plus adaptées, plus justes et plus transparentes, au bénéfice des élus et des sinistrés de nos territoires.

en 2021, à l’occasion d’un déplacement en Corrèze, le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin avait annoncé que des agents d’administration centrale en poste en Île de France seraient redéployés dans des villes se portant candidates pour les accueillir. Le 16 mars 2022, il communiquait le nom des vingt retenues, parmi lesquelles figurait Cahors, appelée à recevoir, en centre ville, une antenne de l’inspection générale de la gendarmerie nationale En tant que maire, j’avais salué cette initiative qui renforçait le lien de proximité entre l’action publique et les Français, offrait une opportunité de développement aux territoires et répondait à l’aspiration de nombreux agents de travailler dans un autre cadre de vie. La relocalisation de ce service a été programmée à l’horizon 2025. Le chef de I’IGGN s’est récemment rendu à Cahors pour évoquer les modalités concrètes d’installation des trente deux agents concernés. Or des incertitudes semblent désormais peser sur ce redéploiement. J’ai interrogé, le 13 novembre dernier, le directeur général de la gendarmerie nationale : il m’a indiqué que les plans de relocalisation du ministère de l’intérieur sont actuellement remis à l’étude, au regard des coûts importants induits par ces transferts. Un renoncement de la part du Gouvernement serait jugé inacceptable et une telle décision décrédibiliserait les élus qui se sont démenés sur le terrain pour faire aboutir ce projet et qui l’ont publiquement annoncé. Monsieur le secrétaire d’État, pouvez vous me confirmer que l’engagement pris par l’État

leur état nécessite des travaux d’aménagement pour un montant estimé à 1,2 million d’euros. Concernant le logement des militaires, la gendarmerie envisage de procéder à des prises à bail.

ronger les territoires. Le respect de la parole de l’État obéit à un principe de crédibilité et de continuité. Ce principe vaut pour votre gouvernement comme pour celui qui pourrait vous succéder.

à Lyon et dans le département du Rhône. Le ministère de l’intérieur a régulièrement communiqué sur des renforts de policiers et de gendarmes nationaux dans cette circonscription. Dans une optique de bonne coopération entre l’État et les communes,

passées et à venir, en contradiction avec les promesses de Gérald Darmanin. Maintenir la sécurité publique devient de plus en plus difficile. L’opacité sur les effectifs réels est dommageable et pourrait laisser à penser que les renforts annoncés ne seraient en réalité que le remplacement de départs. De telles arrivées ne suffiraient même pas à combler ces derniers, les effectifs globaux étant apparemment en baisse sur la DIPN du Rhône, d’après ces syndicats. Cette situation n’est pas tenable. Aussi, nous souhaitons savoir si le Gouvernement envisage de communiquer le solde net des effectifs de police,

par un cours d’eau et près de 75 % des habitants vivent à moins de deux kilomètres de l’eau. Ce lien entre les Val de Marnais et leur fleuve, autrefois marqué par la baignade et les loisirs aquatiques, reste fort dans les mémoires locales. Le défi est écologique et sanitaire. Pour y répondre, les collectivités locales ont investi, avec l’État, plus de 200 millions d’euros dans des infrastructures de dépollution et d’assainissement.

Cette ambition ne peut se concrétiser sans un soutien fort et durable de l’État. La baignabilité de nos cours d’eau constitue un enjeu majeur pour l’attractivité de nos territoires et pour le bien être de nos concitoyens. Monsieur le ministre, pouvez vous dresser un état des lieux des mesures que votre ministère met en œuvre pour accompagner les élus locaux val de marnais dans leurs efforts d’assainissement ? Comment comptez vous garantir que l’héritage des Jeux profite concrètement et durablement aux habitants en leur offrant un

avec les opérateurs de l’assainissement et les collectivités locales, a réussi à relever ce défi en un temps record, alors que ces chantiers, nombreux et complexes, auraient dû durer des décennies. Le principal héritage du plan sera donc l’ouverture de sites de baignade pérennes dès l’année 2025 sur la Seine et sur la Marne. Pour ce faire, il faut mettre fin au plan initial, notamment résorber les mauvais branchements restants et finir les travaux sur le réseau public de collecte.

puis à l’aval. L’État, au travers de l’agence de l’eau Seine Normandie, subventionne les travaux de correction de mauvais branchements, avec une majoration de 20 % des forfaits d’aide sous maîtrise d’ouvrage publique. Il subventionne également les travaux sur les réseaux d’assainissement, à 60 %, pour améliorer encore la qualité de l’eau. les services de l’État accompagnent chaque collectivité pour la mise en œuvre des procédures réglementaires préalables à l’ouverture des sites de baignade. Nous sommes donc pleinement engagés aux côtés des acteurs concernés pour assurer durablement la baignabilité des eaux et permettre à nos concitoyens d’en profiter pleinement. La parole

de rénovation, faute de savoir si l’État les soutiendra. Interrogés, les services de la préfecture de région nous ont répondu que la réhabilitation de 9 900 900 logements a déjà coûté 124 millions d’euros à l’État, soient 24 millions de plus que l’enveloppe initiale, bénéficiant ainsi à 12 400 foyers. Qu’en est il donc des 13 100

Engagement pour le renouveau du bassin minier, lancé en 2017. À la demande de la ministre Valérie Létard, qui a d’ores et déjà eu l’occasion de le faire au Parlement et hier encore lors de son déplacement à je reprendrai l’historique de manière claire. L’État s’est engagé à cofinancer de 2017 à 2027 un programme de rénovation des cités minières, à hauteur de 100 millions d’euros pour la rénovation des logements et de 100 millions d’euros pour l’aménagement des espaces publics. Sur le volet rénovation, qui concerne le ministère du logement, les financements de l’État atteignent 124 millions d’euros à la fin de 2024. L’engagement initial de 100 millions d’euros de subventions est donc d’ores et déjà dépassé. Comme Valérie Létard s’y est engagée, le Gouvernement ajoutera 8 millions d’euros supplémentaires au budget 2025. Sur le volet espaces publics, qui concerne le ministère chargé des collectivités, l’État aura engagé entre 2022 et la fin de 2024 plus de 42 millions d’euros, soit près de la moitié de l’enveloppe. Il reste encore trois ans d’ici à 2027 pour engager la seconde partie. L’engagement des subventions est donc en ligne avec le calendrier des projets. Concernant la budgétisation de 2025, le ministère des collectivités a confirmé l’engagement de l’État à hauteur de 17,5 millions d’euros,

aucune instance de dialogue entre la maîtrise d’ouvrage et les villes. Malgré des demandes répétées au préfet de région, la municipalité de La Courneuve ne dispose d’aucune d’information claire quant aux modalités d’isolation phonique envisagées. Une étude d’impact de 2004 établissait déjà que ce projet engendrerait des pollutions sonores considérables. Or cette dernière ne prenait pas en compte les développements du territoire engagés depuis vingt ans par la municipalité et son maire, Gilles Poux, dont la nouvelle zone d’aménagement Pour pallier cette carence, la ville a proposé à Plaine Commune de mener une étude acoustique, mais le projet a avorté, faute de retour du maître d’ouvrage. À ce jour, seule une enveloppe de 15 millions d’euros est prévue pour la mise en place de protections acoustiques, soit moins de 1 % du budget global. C’est une somme insuffisante, qui ne permettra d’intervenir que sur la moitié du tracé.

d’aucun des avantages liés à la mise en ligne du Charles de Gaulle Express, mais en subiront toutes les nuisances et les conséquences. Monsieur le ministre, nous vous demandons trois choses. de contraindre à une clarification de l’ensemble des bâtiments de La Courneuve qui doivent faire l’objet de mesures d’isolation, et à une réintégration des bâtiments oubliés depuis l’inventaire de 2018. Deuxièmement, nous vous demandons d’imposer que l’enveloppe dédiée aux protections acoustiques pour la ville de La Courneuve et toutes les autres soit réévaluée et augmentée. d’imposer une concertation renforcée entre la maîtrise d’ouvrage et la ville de La Courneuve. Très bien Express a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en décembre 2008, à la suite de l’enquête publique menée en 2007, et avant la construction de la ZAC de La Courneuve : c’est pourquoi les études d’avant projet ne comprennent pas d’éléments ou de prescriptions relatives à l’atténuation du bruit pour les riverains. En l’espèce, ils n’étaient pas encore riverains de cette nouvelle infrastructure, qui présente

au delà des exigences initiales. Cela a permis de résorber l’ensemble des points noirs « bruits ferroviaires » préexistants au projet. Au delà des écrans acoustiques retenus lors de l’enquête publique, qui permettront une réduction du bruit à la source, des travaux pour améliorer la performance acoustique des façades des bâtiments seront réalisés afin de protéger les riverains à l’intérieur des habitations. Les diagnostics sont en cours pour permettre la réalisation de ces travaux qui se concentreront en particulier

d’un véritable statut de l’élu local, sollicité par tous depuis de très nombreuses années. Depuis le dernier renouvellement municipal, nous assistons à un véritable « blues des maires » et nombreux sont ceux à avoir raccroché l’écharpe. Depuis 2020, 2 400 maires ont démissionné et 57 000 sièges de conseiller municipal sont vacants. Confrontés à toujours plus de normes, de contraintes, mais aussi de responsabilités, les élus locaux nous font remonter un sentiment de découragement et de solitude. Figures

Il est indispensable d’inciter les concitoyens à continuer à s’engager et à prendre des responsabilités au sein de nos communes. Ma question est donc simple, même si j’imagine que la réponse est complexe au regard du contexte politique : à quand un véritable statut de l’élu local dans notre pays ? La parole est à M. le ministre

transmettre quelques éléments d’éclairage. Le Gouvernement partage évidemment l’objectif d’améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux, notamment dans la perspective des élections municipales de 2026. Il s’emploie d’ores et déjà à soutenir l’ensemble des élus dans l’exercice de leurs missions. Ce soutien s’est notamment traduit par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui a introduit de nombreuses dispositions visant à accompagner les élus locaux, notamment des communes rurales, dans l’exercice de leur mandat – je pense, par exemple, à la revalorisation des indemnités de ces élus ruraux. Par ailleurs, afin de faire face à la hausse des violences commises à l’encontre de personnes titulaires d’un mandat électif, le Gouvernement a soutenu l’adoption de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Cette loi a notamment alourdi les sanctions pénales encourues par les auteurs de violences faites aux élus et a prévu un dispositif d’octroi automatique de la protection fonctionnelle pour les exécutifs locaux. Enfin, dans le prolongement des différents travaux que vous évoquez, qu’il s’agisse des rapports parlementaires ou de la convention nationale pour la démocratie locale organisée par le Gouvernement le 7 novembre 2023, de nombreuses réflexions ont été menées et ont trouvé une traduction dans la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local, sur l’initiative des sénateurs Bruno Retailleau, François Noël Buffet, Françoise Gatel, Mathieu Darnaud et Hervé Marseille. Comme cela par le Premier ministre lors de la clôture du Congrès des maires, cette proposition de loi, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 7 mars 2024, sera examinée par l’Assemblée nationale en février 2025 si le contexte particulier que vous avez évoqué le permet. À cette occasion, et en y intégrant le produit des échanges très constructifs qui se sont poursuivis avec les associations d’élus locaux, Catherine Vautrin proposera de l’enrichir de dispositions complémentaires destinées à faciliter l’exercice du mandat d’élu local et à le protéger. décentralisation. Monsieur le ministre, comme vous, j’ai assisté aux Assises des départements de France. Nos départements sont en sursis. Conseillère départementale de la Vienne, je constate un effet de ciseaux significatif en fonctionnement, à titre onéreux (DMTO) de 23 millions d’euros entre 2022 et 2024 et, dans le même temps, une augmentation des dépenses supplémentaires imposées par l’État, non ou mal compensées, à hauteur de 23 millions d’euros, soit une perte de 46 millions d’euros en trois ans. À cela s’ajoutent l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. Pourtant, le projet de loi de finances exige un nouvel effort susceptible de mettre « en impasse budgétaire » près de 85 % des départements d’ici à la fin de 2025. Pour la Vienne, c’est 16 millions d’euros d’économies à réaliser. Nous sommes dans une impasse financière, avec cette particularité que les dépenses des départements ne sont pas pilotables. Comme vous, j’ai écouté attentivement le discours du Premier ministre. Je partage son constat : le modèle départemental que nous connaissons a atteint ses limites. Je partage également son souhait « d’inventer un autre modèle » pour mener à bien les projets Maintenant que cela est dit, qu’allez vous faire ? Nos départements sont en première ligne pour accompagner la ruralité et les populations fragiles face aux défis du bien vieillir et aux enjeux de sécurité civile. civile. Quelle commune allons nous cesser d’accompagner ? Quelles routes, quel patrimoine allons nous cesser d’entretenir ? Quelle population du département allons nous devoir abandonner ? Si rien n’est fait, au printemps prochain, trente départements, dont la Vienne, n’auront d’autre choix que de vous remettre leurs clés. La mise en œuvre du 49.3 et le dépôt de motions de censure compliquent évidemment la donne. Je souhaite que le Gouvernement soit confirmé pour que nous puissions avancer et répondre aux attentes nombreuses des Français. Si tel était le cas, donnerez vous suite aux propositions de Départements de France

Premier ministre a eu l’occasion de rappeler à la fois son soutien aux élus, sa connaissance de la difficulté des départements et sa volonté de réduire de manière significative le niveau d’efforts demandés aux collectivités. Qu’il me soit permis de saluer l’esprit de responsabilité qui a animé les présidents de département et les conseillers départementaux

le taux de DMTO pendant une période de trois ans. Sur la base d’une estimation de 2024, cela pourrait générer de l’ordre de 1 milliard d’euros de recettes supplémentaires. Le Gouvernement a également entendu travailler

Lille. La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) s’inquiète de la qualité de l’offre et du manque de fiabilité des liaisons Intercités. Le nombre de voyages sur la liaison Intercités Nantes Bordeaux a crû de 90 % entre 2019 et 2022, avec le passage de trois à quatre allers retours par jour depuis 2021.

De plus, le service est dégradé par un tronçon en voie unique sur Nantes Bordeaux et une signalisation obsolète, ainsi que par des limitations de vitesse dont la cause est la vétusté des voies. Pour satisfaire la demande, le parc roulant doit se développer et proposer davantage de convois à deux rames accolées. Suivant les attentes des usagers, un quatrième aller retour Nantes Lyon est il envisagé ?

Le dynamisme démographique de la Loire Atlantique et de la région Pays de la Loire plaide sérieusement pour un renforcement de l’offre ferroviaire sur l’arc Atlantique. La

pour restaurer les performances de vitesse nominale et augmenter les capacités, notamment sur La Rochelle Saintes Bordeaux. Le réseau ferré de la ligne Nantes Lyon fera également l’objet de travaux de rénovation en 2027 pour supprimer les limitations de vitesse, notamment sur la section Bourges Saincaize.

que traverse le territoire de la Camargue, où l’exposition au risque d’inondation menace gravement la sécurité de 30 000 habitants et celle de 200 000 personnes supplémentaires en période touristique. Après les crues désastreuses de 1993, de 1994 et de 2003, le plan Rhône a été mis en place, sous l’égide de l’État, pour protéger les populations riveraines en améliorant les digues. Depuis lors, 220 millions d’euros ont été investis et 73 kilomètres de digues ont été renforcés. Cependant, la Camargue gardoise, la Camargue insulaire et la plaine de Beaucaire restent aussi vulnérables qu’il y a vingt ans. Le syndicat mixte interrégional Symadrem a déposé, en avril 2022, une demande d’autorisation environnementale pour des travaux essentiels sur les digues du Petit Rhône. Ce projet, en parfaite conformité avec le plan Rhône et le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022 2027, permettrait de protéger efficacement ces zones sensibles, tout en préservant l’équilibre environnemental et agricole du territoire. Malgré les engagements pris dans le contrat de plan interrégional État région Rhône Saône 2021 2027, cette demande d’autorisation est actuellement suspendue. Le temps presse, nous devons éviter de nouvelles tragédies comme celles de 2003, d’autant que les élus de la Camargue ont, depuis vingt ans, soutenu les travaux en amont, sans bénéficier eux mêmes des protections qu’ils ont contribué à financer. je vous demande de tout mettre en œuvre pour lever cette suspension et permettre la mise en enquête publique de ce dossier afin de garantir le démarrage des travaux dès 2025. L’État ne doit pas tourner le dos aux engagements pris envers la Camargue et ses habitants.

dans la protection de la Camargue aux côtés de ses élus, sous réserve que ce projet prenne en compte les enjeux spécifiques du territoire, notamment la sécurité de ses habitants lors des crues, la réduction des potentiels dommages, la préservation de la biodiversité, le maintien de l’agriculture, ce qui suppose de limiter la salinisation des sols, en partie par des apports d’eau douce pendant les crues du fleuve. Une étude menée par les services de l’État a confirmé la nécessité, pour le secteur amont du Petit Rhône, de sécuriser en priorité les huit premiers kilomètres de digues, tant en rive gauche qu’en rive droite, pour protéger le secteur très urbanisé de Trinquetaille à Arles ainsi que la plaine de Fourques. Elle a également mis en avant des solutions alternatives

prévention des risques. Monsieur le ministre, depuis son annonce en 2022, le projet d’installation de stockage des déchets dangereux (ISDD) d’Hersin Coupigny, dans le Pas de Calais, suscite l’inquiétude générale sur le territoire. Le 18 octobre 2024, le groupe Veolia et sa filiale Sarpi Mineral France ont déposé une demande d’autorisation environnementale auprès de la préfecture afin de créer cette zone de stockage. Depuis trois ans, les élus des communes directement concernées s’opposent à ce projet, tout comme le conseil départemental et le conseil régional. L’inquiétude est

L’incompréhension s’ajoute à l’inquiétude, le projet prévoyant le stockage de déchets dangereux issus d’autres régions qui représentent un quart du territoire de la France métropolitaine. Enfin, ce projet cumule des effets délétères pour les conditions de vie et de santé de la population, mais aussi en termes de protection de la nature et de la biodiversité, en particulier pour le parc départemental voisin

de stockage des déchets dangereux sont des équipements importants pour la protection de l’environnement : elles permettent de ne pas disperser dans le milieu naturel les polluants que ces déchets contiennent. Pour un certain nombre de déchets dangereux, il s’agit de la seule solution de traitement adaptée pour les éliminer en toute sécurité. Dans ce contexte, les législations européenne et française prévoient que l’implantation de ce type d’installation respecte le principe de proximité. En d’autres termes, chaque région doit être la plus autonome possible pour gérer les déchets produits sur son territoire et éviter de les exporter vers une région voisine. Dans les Hauts de France, il n’existe plus d’installation de stockage des déchets dangereux depuis la fermeture du site de Menneville en 1994. Les déchets dangereux de la région sont donc actuellement transférés vers des régions voisines, en contradiction avec ce principe de proximité. S’agissant de ce projet S’agissant de ce projet d’ISDD, une phase d’échanges avec les acteurs locaux et les habitants a débuté il y a plus de deux ans. Une concertation préalable s’est déjà tenue à l’automne 2022, sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). Celle ci a permis à l’exploitant d’améliorer son projet pour tenir compte de certaines recommandations. Pour répondre aux craintes que vous évoquez, soyez assurés que les services de l’État chargés de l’instruction de ce dossier seront vigilants à ce que les conditions de stockage garantissent un niveau de protection de l’environnement le plus élevé possible.

non collectif (ANC) aux communes de moins de 200 habitants. Cela exclut de nombreux petits villages, comme Champguyon – 290 habitants – ou Neuvy – 271 habitants. Bien que ce seuil vise probablement à cibler les communautés les plus modestes, il prive les habitants de communes légèrement plus grandes, mais tout aussi rurales et aux ressources limitées, du soutien nécessaire pour se conformer aux normes environnementales actuelles. L’assainissement individuel représente un investissement important et beaucoup d’habitants de petites communes peinent à financer ces mises aux normes. Il serait donc opportun que cette subvention soit élargie à toutes les petites communes, ce qui permettrait à des milliers de foyers dans des situations similaires d’améliorer leurs installations. Cela contribuerait également à préserver la qualité de l’eau et l’environnement, des objectifs essentiels que nous partageons tous. Étant donné que l’agence de l’eau est un établissement public sous la tutelle du ministère de la transition écologique, entendez vous revoir les critères d’éligibilité pour permettre aux petites communes, notamment rurales,

dans des communes pour lesquelles des prescriptions de réhabilitation d’assainissement non collectif sont identifiées à l’issue des profils de vulnérabilité des zones de baignade intérieures et dans un arrêté de déclaration d’utilité publique (DUP) de protection de captage pour l’alimentation en eau potable. Troisièmement, il doit

porte sur le projet d’arrêté cadre fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans. Dans l’Ain, les étangs de la Dombes forment un ensemble unique qui associe la production piscicole à une biodiversité singulière. Ainsi la filière piscicole est une activité emblématique du territoire qui s’inscrit dans la préservation du patrimoine naturel. À la lecture du projet d’arrêté ministériel mis en consultation, relatif à la gestion des populations de cormorans, les professionnels aindinois de la pisciculture constatent avec amertume qu’il n’a pas été tenu compte des discussions qui se sont tenues sur le contenu dudit projet. projet. Les modifications qui sont aujourd’hui envisagées marqueraient un retour en arrière important, annihileraient le travail fructueux qui a été engagé pour le territoire et menaceraient l’équilibre de l’écosystème local. L’adoption en l’état de l’arrêté serait notamment en totale contradiction avec la note stratégique de la fin de 2023 du Haut Commissariat au plan qui présente le développement de l’aquaculture comme un enjeu de souveraineté alimentaire.

extensive en étang continental, qui ont à cœur d’assurer une production qualitative tout en préservant la biodiversité associée aux milieux

qu’un certain nombre de partenaires ont fait parvenir aux services d’Agnès Pannier Runacher leurs remarques et propositions d’évolution sur l’arrêté que vous avez évoqué. Celui ci a fait l’objet d’une consultation du Conseil national de la protection de la nature le 16 octobre dernier, puis d’une consultation publique du 18 octobre au 8 novembre. À l’issue de cette consultation du public, qui s’est révélée favorable au projet d’arrêté proposé, les échanges se sont poursuivis avec les partenaires. Une réunion bipartite avec les représentants des pisciculteurs a ainsi été organisée le 14 novembre dernier afin de discuter de nouvelles évolutions possibles du texte. du texte. Postérieurement à cet échange, de nouvelles contributions des représentants des pisciculteurs sont parvenues aux services de la ministre le 19 novembre et ont fait l’objet d’une analyse attentive.

sur notre pisciculture, mais également sur les espèces protégées de nos rivières. Les évolutions envisagées portent sur un meilleur suivi des destructions, un encadrement des dérogations sur les eaux libres, un aménagement de la période de destruction

vous n’êtes pas sans savoir que les porteurs de projets éoliens terrestres ont l’obligation de respecter des normes acoustiques définies aux articles 26 et 28 de l’arrêté du 26 août 2011. Or il se trouve que de récentes décisions judiciaires ont condamné des promoteurs, pourtant en règle à l’égard des protocoles de mesure, retenant que le respect des normes prônées par ces protocoles ne garantissait pas efficacement la santé et la sécurité du voisinage, expressément visées dans notre droit. En effet, les basses et très basses fréquences, ainsi que les modulations d’amplitude, qui sont pourtant à la source des troubles ayant conduit à ces condamnations, sont toujours ignorées, par dérogation à l’encadrement des nuisances sonores prévues par le code de la santé publique.

par les projets éoliens terrestres, au regard de critères liés à l’intensité des nuisances et à la répétition des bruits. Le dernier protocole de mesure du bruit élaboré par le Gouvernement, entré en vigueur en 2021, annulé par le Conseil d’État pour défaut d’évaluation environnementale en mars dernier, n’intégrait d’ailleurs toujours pas ces critères. Ma question est simple, monsieur le ministre. Puisque la réglementation en vigueur est, insuffisante et préjudiciable, quand et comment comptez vous garantir rapidement la prise en compte des impératifs de santé pour les riverains, qui sont de plus en plus nombreux, dans les instruments de mesure des nuisances sonores provoquées par les installations éoliennes terrestres ? La

pour de nombreux Français et peuvent avoir un effet majeur sur la santé publique. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a lancé ces dernières années de nombreuses actions pour réduire le bruit, notamment celui des éoliennes. Avant toute autorisation d’un parc éolien, une étude d’impact est déposée, une étude acoustique. Depuis 2021, un contrôle acoustique systématique a lieu dans les douze mois suivant la mise en service des parcs éoliens.

les seuils ni la validité des méthodes proposées. Le rapport que vous mentionnez a justement permis de constater que les mises à jour des protocoles acoustiques en 2022 ont amélioré

parcs éoliens, qui sont nécessaires à la transition énergétique et aux objectifs de décarbonation du pays, se fasse en bonne intelligence avec les populations riveraines. Celles ci ne doivent en aucun cas

chargée de l’énergie. Monsieur le ministre, j’attire votre attention sur une question qui touche au cœur de nos territoires, à leur identité et à leur patrimoine : l’impact des éoliennes sur nos paysages historiques, qui font la renommée et l’attractivité de nos communes rurales et de nos campagnes. Face à ces transformations, certains producteurs et exploitants d’énergies renouvelables dans le domaine éolien proposent des dispositifs de chèque énergie à destination des résidents des communes qui accueillent ces installations. Si l’intention semble louable – il s’agit de redistribuer une partie des bénéfices et de favoriser l’acceptation locale cette pratique soulève des questions fondamentales. D’abord, d’un point de vue juridique, ces initiatives sont elles conformes au droit français ? Peuvent elles être interprétées comme des contreparties directes, voire des mécanismes visant à compenser l’impact de ces projets sur des paysages, qui, je le répète, constituent un élément indissociable de notre patrimoine national ? Ces paysages, façonnés par des siècles d’histoire, sont bien plus que de simples espaces ruraux : ils sont le reflet de nos racines, de notre culture, et un atout majeur pour le tourisme et la vie locale. Leur transformation par les éoliennes, parfois imposées sans réelle concertation, donne souvent un sentiment d’impuissance à nos concitoyens. Ces chèques, bien qu’ils soient apparemment bénéfiques, ne risquent ils pas de masquer un problème plus grave : la destruction progressive de nos horizons ? Est il acceptable que la réponse soit laissée à des initiatives privées, sans un cadre clair et national qui garantirait une gestion équilibrée et respectueuse de nos territoires ? Enfin, ne serait il pas nécessaire d’évaluer ces dispositifs à l’aune de leur équité entre communes et de leur véritable impact ? Une telle compensation ne devrait elle pas relever d’un mécanisme institutionnel plus transparent et plus adapté, qui prendrait en compte l’intérêt général, la protection du patrimoine et la transition énergétique ? Monsieur le ministre, quelles mesures le Gouvernement entend il prendre pour assurer que la transition énergétique, qui est indispensable, ne se fasse pas au détriment de nos paysages et de l’identité de nos territoires ? La parole est à M. le ministre M. le ministre délégué. Monsieur le sénateur, je connais votre sensibilité sur le sujet des éoliennes, particulièrement dans votre région. Vous m’interrogez sur la légalité d’un chèque énergie mis en place par les producteurs et exploitants des énergies renouvelables à destination des résidents des communes accueillant des éoliennes. éoliennes. Je précise que le chèque énergie qui existe aujourd’hui est une aide de l’État à destination des ménages les plus modestes, afin de les aider à payer leurs factures d’énergie, sans aucun lien géographique. Ce que vous évoquez est un autre outil,

l’acceptabilité du déploiement des énergies renouvelables, un gain financier pour les territoires d’accueil, ce qui n’exclut évidemment pas d’autres considérations environnementales auxquelles vous êtes particulièrement sensible. Agnès Pannier Runacher me charge de vous dire qu’elle est tout à fait disposée à retravailler avec vous sur ce dispositif.

Si l’objectif de sobriété foncière est justifié, sur le terrain, de nombreuses difficultés juridiques et pratiques découlent de sa mise en œuvre. Face aux difficultés rencontrées par les élus,

mois après le vote de la loi, envisagez vous de publier rapidement le décret relatif au mécanisme de la garantie rurale, prévoyant qu’une commune ne peut se voir attribuer d’ici à 2031 une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers inférieure à 1 hectare dès lors qu’elle est couverte par un document d’urbanisme

par an, en moyenne, dans notre pays. L’impératif de sobriété foncière est une responsabilité commune, dont la mise en œuvre doit évidemment être différenciée. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit une trajectoire progressive et une modulation de l’objectif selon les spécificités de chaque territoire. La construction dans les communes n’est pas bloquée. Les schémas régionaux, ainsi que les documents de planification et d’urbanisme, permettent aux collectivités territoriales de moduler l’objectif selon leurs besoins et leurs spécificités. Par ailleurs, la loi prévoit que toute commune couverte par un document d’urbanisme antérieur à août 2026 ne peut être privée d’un potentiel minimum

si nécessaire. Pour terminer, je vous rappelle que le Premier ministre Michel Barnier a indiqué sa volonté de revoir les conditions du zéro artificialisation nette. J’espère que la période que nous vivons aujourd’hui permettra d’atteindre l’objectif bien compris que vous avez relayé dans cette assemblée.

Le Gouvernement est mobilisé aux côtés des élus et le ministère de la justice s’investit pleinement dans la lutte engagée contre ces atteintes, quelle que soit la forme qu’elles sont susceptibles de revêtir.

diffusée le 3 juillet 2023 et à la préparation de laquelle le ministère de la justice a naturellement pris part. L’action du ministère de la justice est, depuis plusieurs années déjà, pleinement cohérente avec les objectifs et actions de ce plan national. Ce sujet d’importance a fait l’objet, ces dernières années, de plusieurs circulaires tendant à permettre aux parquets de répondre de manière ferme et cohérente aux atteintes aux élus portées à leur connaissance et à mieux accompagner ces derniers lorsqu’ils sont victimes. Cette action doit être poursuivie et renforcée. La loi du 21 mars dernier renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a permis d’élargir le spectre des atteintes aux élus, en y incluant de façon pertinente les candidats aux élections, en aggravant certains niveaux de peine ou en parachevant les mécanismes juridiques d’information des élus. La réponse pénale, à cet égard, est ferme et doit le rester. Ainsi que le garde des sceaux l’a récemment dit dans cet hémicycle, il aura l’occasion de le rappeler aux procureurs généraux. Récemment, la Chancellerie a aussi rappelé les outils à la disposition des juridictions et mobilisé l’ensemble de la chaîne pénale. Elle a également adressé aux procureurs généraux un modèle de protocole relatif au renforcement des relations entre les parquets et les maires. Le garde des sceaux entend aujourd’hui évaluer l’efficacité de ces évolutions normatives en s’assurant de la pertinence du cadre juridique mis en place. Il compte notamment réunir à intervalles réguliers les référents dédiés aux atteintes aux élus pour que les remontées de terrain nourrissent notre réflexion collective.

en troisième position derrière Chypre et la Roumanie. On le sait, la politique carcérale en France consiste à construire de nouveaux établissements pénitentiaires. À Gradignan, en Gironde, le nouveau bâtiment tant attendu a été livré

a annoncé un plan anti drones très prochainement. Pouvez vous nous donner des éléments sur ce plan, de manière que l’on puisse rassurer les surveillants pénitentiaires ? La parole Mme la secrétaire d’État. Le garde des sceaux vous remercie, madame la sénatrice, de votre question, qui permet d’aborder la situation complexe dans laquelle nos prisons se trouvent aujourd’hui et le plan spécifique déjà mis en œuvre par le Gouvernement pour y apporter des solutions pérennes et efficaces et lutter contre la surpopulation carcérale. carcérale. Les travaux de reconstruction du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan ont démarré en 2021 et sont organisés en deux grandes phases d’aménagement, de manière à assurer la continuité de l’activité de l’établissement existant. Ce projet répond à plusieurs ambitions : d’une part, améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires, permettre une meilleure prise en charge des personnes détenues et améliorer l’accueil des partenaires ; d’autre part, assurer une meilleure intégration de l’établissement dans la cité. Le coût total prévisionnel de cette reconstruction s’élève à environ 183 millions d’euros. La livraison des nouveaux bâtiments de l’établissement a eu lieu le 20 mai 2024. Toutefois, il s’agit seulement de la première phase du projet. La seconde phase doit notamment permettre de perfectionner les travaux déjà réalisés et d’installer de nouveaux équipements de sécurité. En effet, le centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan a déjà été livré d’un dispositif anti drones. Les travaux de câblage sont en cours et la mise en service est programmée très prochainement. pénitentiaire figure également sur la liste des établissements identifiés comme étant prioritaires au titre de l’année 2025 pour la dotation des dispositifs de brouillage de communications illicites. La modification du système de caillebotis pour renforcer les fenêtres, qui autorise désormais le démontage du vitrage pour son remplacement en cas de bris, est également à l’étude, pour une réalisation prévue durant la seconde phase des travaux. La parole

Comme vous le rappelez, en l’état de la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil, les seuls signes diacritiques autorisés dans la langue française sont les points, trémas, accents et cédilles. L’Académie française, sollicitée en 2014, a confirmé qu’il s’agissait des seuls signes diacritiques propres à la langue française. Le tilde n’en fait donc pas partie. Il est exact que, en février 2019, lors de la signature du contrat d’action publique pour la Bretagne, l’un des engagements du Premier ministre portait sur l’ouverture d’une réflexion sur les conditions d’intégration à l’état civil de tels signes régionaux. Une étude a été engagée par le ministère de la justice afin de recenser l’ensemble des adaptations rendues nécessaires par une telle intégration. Celle ci a été envisagée à l’article 9 de la loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, qui prévoyait d’autoriser les signes diacritiques des langues régionales dans les actes de l’état civil. Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mai 2021, a censuré cette disposition au titre de l’article 2 de la Constitution, qui énonce que « la langue de la République est le français ».

Nos forces de sécurité méritent, bien sûr, notre attention de tous les instants. C’est vrai en particulier de nos sapeurs pompiers, exposés aux incendies. En effet, rappelons que, lorsque les gens fuient pour échapper à la fumée, nos soldats du feu y pénètrent.

les tableaux de maladies professionnelles, soit en les révisant, soit en en créant de nouveaux, afin de mieux accompagner nos sapeurs pompiers dans cette épreuve. C’est une priorité pour eux ; c’est un devoir pour nous. La parole est à Mme la secrétaire

d’abord, du fait de son exposition potentielle aux fumées de combustion, la profession bénéficie des mesures de prévention prévues par le code du travail relatives aux expositions aux agents chimiques, qui visent notamment à minimiser les expositions à un niveau aussi bas que techniquement possible et à renforcer la surveillance médicale. Concernant la réparation des pathologies professionnelles, comme vous le soulignez, les tableaux de maladies professionnelles n 43 et 45 mentionnent explicitement les travaux d’extinction des incendies pour la réparation du carcinome du nasopharynx et les services de secours et de sécurité pour celle du carcinome hépatocellulaire. Par conséquent, les pompiers peuvent déjà bénéficier d’une reconnaissance automatique de maladie professionnelle pour ces deux pathologies. Par ailleurs, sur saisine du ministère du travail, l’Anses a publié un rapport en octobre 2024 dans lequel elle fait état d’un niveau de corrélation avéré entre les cancers de la vessie, de la plèvre ou du péritoine et la profession de pompier. À noter que ces pathologies figurent respectivement dans trois tableaux des maladies professionnelles. Ainsi, pour les pompiers relevant du régime de droit privé, la reconnaissance devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est donc déjà possible. Compte tenu du fait que les tableaux de maladies professionnelles s’imposent à l’ensemble des régimes, le ministère chargé du travail a entamé les démarches nécessaires à leur révision

des Français de l’étranger. Madame la ministre, dès le 8 octobre 2023, les résidents du nord de l’État d’Israël ont été évacués par le gouvernement israélien, à la suite des bombardements du Hezbollah. Jusqu’à présent, ils n’ont pas été en mesure de revenir chez eux. Si un cessez le feu a enfin pu être prononcé, la situation reste fragile, comme on l’a vu ces derniers jours. Parmi ces résidents se trouvent des centaines de familles françaises. Nos autorités consulaires ont réalisé un important travail de recensement et de soutien de ces familles, qui n’étaient que partiellement inscrites au registre des Français établis hors de France, ce qui a rendu leur repérage Serait il possible de nous éclairer sur le bilan de cette opération et de savoir combien de personnes ont été recensées ou aidées ? Combien continuent à être suivies aujourd’hui et dans quelle mesure ?

au gré des mouvements de nos différentes lignes diplomatiques. La parole

qui résident en Israël et qui sont touchées par la situation sécuritaire. Cela vaut, d’ailleurs, au nord comme au sud du pays. Ces familles n’ont pas encore pu rentrer chez elles, mais nous espérons que le cessez le feu le feu intervenu le 26 novembre entre Israël et le Liban permettra le retour sûr des déplacés. Vous l’avez dit, nos services consulaires ont réalisé un important travail de recensement de ces familles, qui représentent 5 000 personnes dans le nord d’Israël et 6 000 à la frontière de la bande de Gaza. Le ministère a immédiatement consenti un effort budgétaire pour les soutenir, d’abord en abondant de 50 000 euros l’enveloppe de secours occasionnel du consulat général à Tel Aviv.

du nord d’Israël (AFSNI) et au club des Français d’Ashkelon, qui sont eux venus en aide à des centaines de familles. Nos services ont également été mobilisés pour fournir aux familles, dès octobre 2023, un soutien consulaire

J’attire l’attention de Mme la ministre de la santé et de l’accès aux soins sur le fonctionnement des pharmacies à usage intérieur (PUI) en milieu rural. Les PUI répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge au sein des établissements de santé, de certains établissements médico sociaux ou encore par les services d’incendie et de secours. Leur rôle est essentiel dans la qualité et la sécurité du

Je vous remercie, Comme vous le rappelez, les pharmacies à usage intérieur jouent un rôle essentiel dans la qualité et la sécurité du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles au sein des établissements de santé, de certains établissements médico sociaux et des services d’incendie et de secours. C’est pourquoi le problème de la démographie pharmaceutique, notamment en établissement de santé, est un sujet de préoccupation majeur, qui nous a conduits à prendre des mesures fortes ces dernières années. Ainsi, depuis 2022, le nombre de postes ouverts pour le diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière est en constante augmentation il est passé de 338 pour l’année universitaire 2022 2023, à 401 pour l’année 2023 2024 et à 441 pour l’année 2024 2025. À moyen terme, ces dispositions devraient permettre de pallier les difficultés de recrutement dans les PUI. Des efforts restent à fournir. Le ministère de la santé et ses services le mesurent et sont très investis en ce sens, afin de permettre aux PUI de continuer à fonctionner. Cela doit se faire sans remettre en cause l’exigence du diplôme de pharmacien hospitalier, garantie de qualité souhaitée par les professionnels et les établissements. Ainsi, des réflexions sont en cours pour renforcer les coopérations et les mutualisations entre les différents établissements de santé et médico sociaux disposant d’une autorisation de PUI. Notre volonté, qui est partagée par les acteurs concernés, est d’améliorer les conditions d’exercice des pharmaciens en PUI en favorisant les coopérations interétablissements.

Le 10 octobre 2024, la Haute Autorité de santé (HAS) a refusé d’accorder une autorisation d’accès précoce à l’un des principaux traitements, le Qalsody, qui vise à ralentir, voire à stabiliser la SLA SOD1, une forme rare de cette maladie.

Ils sont pourtant les plus à même de dire si ce traitement fonctionne ou non face à cette pathologie neurologique évolutive. Dans le département de la Loire, une patiente qui a suivi ce traitement depuis le diagnostic de cette maladie, sur les conseils avisés d’une équipe médicale, a constaté une réelle stabilisation de son état. Plusieurs résultats médicaux permettent de démontrer scientifiquement cette stabilisation depuis la mise en place de ce traitement, qui est approuvé par l’Agence européenne des médicaments depuis le 22 février 2024. Et les exemples ne manquent pas dans d’autres départements… Alors que nous avons ici même adopté une proposition de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies évolutives graves, grâce au courage de notre collègue sénateur Gilbert Bouchet, ces deux avis semblent aller totalement à contresens et poussent les patients à trouver des solutions pour payer un traitement coûtant plus de 30 000 euros. C’est malheureusement une question de vie ou de mort pour eux. Madame la secrétaire d’État, j’ai écrit à ce sujet au Premier ministre le 30 octobre dernier. Il n’est aujourd’hui plus possible d’attendre, pour tous les patients atteints de cette terrible maladie.

Ce dernier a donc pour obligation, post AMM, de fournir des données d’efficacité et de sécurité à plus long terme, d’ici au 30 septembre 2025. septembre 2025. Sur la demande d’autorisation d’accès précoce, la commission de la transparence de la HAS a prononcé un avis défavorable, considérant que les résultats de l’étude comparative placebo, portés au dossier, ne démontraient pas une efficacité statistiquement significative sur le critère de jugement principal. Elle a ainsi émis un refus d’autorisation d’accès précoce pour le Qalsody dans l’attente des données complémentaires post AMM. Considérant le caractère grave et rare de cette maladie, pour laquelle il n’existe pas de traitement approprié,

pour les patients actuellement traités. Au vu de l’AMM octroyée dans cette indication et des rapports de synthèse portant sur vingt huit patients traités dans ce cadre depuis 2022, les autorités sanitaires garantiront aussi la poursuite des initiations de traitement dans l’attente de données complémentaires communiquées par le laboratoire d’ici au 30 septembre 2025.

Pourtant, à l’occasion des jeux Olympiques de Paris 2024, l’activité physique et sportive a été élevée au rang de grande cause nationale… Force est de le constater : au grand dam de bon nombre de spécialistes, de pratiquants et de passionnés, le sport reste un angle mort de nos politiques publiques. Pourquoi est il aujourd’hui nécessaire de reconnaître cette pratique médicale comme telle ? Tout d’abord, la transformation de cette compétence en spécialité serait le vecteur d’une rationalisation de la profession.

de l’activité physique et sportive quotidienne à tous. Vous attirez aujourd’hui notre attention sur la reconnaissance de la médecine du sport en tant que nouvelle spécialité médicale. En France, elle est intégrée dans un cadre dual. D’une part, la médecine du sport est une composante essentielle de la médecine physique et de réadaptation, une spécialité médicale reconnue. Les futurs médecins spécialisés sont ainsi formés à accompagner les patients dans leur parcours de soins, qu’il s’agisse de réhabilitation ou de reconditionnement à l’effort physique. D’autre part, la médecine du sport est une formation spécialisée transversale qui permet par exemple à des étudiants en médecine générale, en rhumatologie ou encore en cardiologie d’acquérir des connaissances et des compétences spécifiques transverses pour répondre aux besoins des patients sportifs. Ce modèle favorise une approche holistique, intégrant la pratique sportive dans une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Comme dans d’autres domaines transversaux, une filière hospitalo universitaire peut se construire sans qu’il existe pour autant un diplôme d’études spécialisées. La création d’une spécialité pourrait fragmenter la prise en charge globale des patients et réduire l’intégration des compétences en médecine du sport au sein d’autres spécialités. En outre, la multiplication des spécialités n’est pas toujours bénéfique pour le système de santé et l’accès aux soins. C’est pourquoi nous avons fait le choix de privilégier une approche mixte, garantissant à la fois la formation spécifique et l’intégration transversale de la médecine du sport, afin de permettre une prise en charge adaptée et globale. Le ministère de la santé et ses services restent toutefois très attentifs aux évolutions des besoins et à leur implication pour la formation. La parole

de l’accès aux soins. Madame la secrétaire d’État, je souhaite vous alerter sur la situation de l’hôpital Édouard Toulouse de Marseille, dont les unités de soins psychiatriques sont les seules à prendre en charge les malades des quartiers nord. Vous le savez, ces derniers comptent parmi les plus pauvres de France et souffrent d’une pénurie chronique de soins spécialisés. Les besoins y sont donc criants. Pourtant, une unité d’admission de l’hôpital Édouard Toulouse a fermé. Ce devait être provisoire, mais les personnels ont la triste habitude de ce qu’ils appellent « le provisoire qui dure ». Cet humour du désespoir cache une réalité devenue insoutenable.

Vous concevrez aisément que privilégier l’ambulatoire n’est pas adapté dans des cités auxquelles il est difficile d’accéder. Faire sortir des patients non stabilisés crée une rupture de soins préjudiciable. ils courent le risque d’une crise, voire d’un passage à l’acte violent, ce qui alimente tragiquement les faits divers. C’est toute la société que le démantèlement des services de soins en psychiatrie met en danger. Cette situation est pour le moins paradoxale, alors que le Premier ministre a dit, ici même, ériger la santé mentale en grande cause nationale de l’année 2025. Dans ce contexte, comment maintenir à Édouard Toulouse une unité de soins psychiatriques essentielle aux habitants ? Comment renforcer encore ses moyens humains et matériels ? La parole est à Mme secrétaire d’État. Madame la sénatrice, le centre hospitalier psychiatrique Édouard Toulouse connaît en effet, comme d’autres structures et depuis plusieurs années, des problèmes importants de recrutement médical et paramédical. Cette situation a conduit sa direction à prendre des mesures provisoires de fermeture de lits du pôle Littoral Nord et de redéploiement des moyens pour garantir une sécurité et une continuité des soins. Ainsi, douze lits ont été temporairement fermés sur les 222 lits d’hospitalisation complète autorisés que compte le centre hospitalier. En parallèle, une unité de soins intersectorielle de vingt quatre lits a été renforcée, de même que les structures extrahospitalières. Enfin, deux lits de crise ont été ouverts. Les équipes de direction sont fortement mobilisées pour recruter des personnels médicaux et rouvrir le plus rapidement possible ces lits d’hospitalisation. Pour y parvenir, l’enjeu est d’assurer l’attractivité de cet établissement auprès des médecins, notamment au travers d’une communication positive à son sujet. Le Gouvernement se mobilise pour accompagner ce type d’établissements à renforcer leur attractivité. Je rappelle par ailleurs que la réforme du financement de la psychiatrie s’est faite avec des moyens supplémentaires,

Sur ce point, même si l’offre de lits souffre d’une pénurie médicale qui la fragilise, on comptabilise, sur le territoire marseillais, près de 160 lits pour 100 000 habitants, ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 80 à 90 lits pour 100 000 habitants. Alpes Côte d’Azur (Paca) demeurent vigilants quant à l’évolution de la situation du centre hospitalier Édouard Toulouse, afin de garantir une réponse aux besoins des patients et une accessibilité aux soins.

La situation de l’hôpital Édouard Toulouse est emblématique. C’est pourquoi, madame la secrétaire d’État, son directeur m’ayant aimablement invitée à visiter son établissement, j’aimerais que vous vous joigniez à nous. La psychiatrie n’est qu’un miroir qui reflète la dégradation des conditions de vie. Il faut donc tout mettre en œuvre pour éviter que des situations déjà tendues ne dégénèrent encore. Nous en La séance est suspendue.